La séance est ouverte. Le compte rendu intégral de la séance du dimanche 25 juillet 2021 a été publié sur le site internet du Sénat. Il n'y a pas d'observation ? Le procès-verbal est adopté. M. le président du Sénat a reçu de M. le Premier ministre communication du décret de M. le Président de la République en date du 1 septembre 2021 portant convocation du Parlement en session extraordinaire à compter du 7 septembre 2021. Acte est donné de cette communication. Ce décret a été publié sur le site internet du Sénat. En conséquence, je constate que la deuxième session extraordinaire de 2020-2021 est ouverte.

cher collègue. Elle sera publiée au et figurera dans l'analyse politique du scrutin. M. Philippe Dallier a fait connaître à la présidence qu'il démissionnait de son mandat de sénateur de la Seine-Saint-Denis à compter du mardi 27 juillet 2021, à minuit. En application de l'article L.O. 320 du code électoral, il a été remplacé par M. Thierry Meignen, dont le mandat de sénateur de la Seine-Saint-Denis a commencé le mercredi 28 juillet, à J'informe le Sénat que, conformément à l'article 8, alinéa 9, de notre règlement, M. Laurent Somon est devenu membre de la délégation sénatoriale aux collectivités territoriales et à la décentralisation le 6 août dernier.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

notre règlement. Monsieur le ministre, mes chers collègues, c'est avec une profonde émotion que nous avons appris le décès, le lundi 30 août dernier, de notre ancien collègue Marcel Henry, qui fut sénateur de Mayotte de 1977 à 2004. La vie et l'engagement de Marcel Henry se confondent avec l'histoire de Mayotte, de son maintien dans la République et de sa transformation en département. Né en 1926, Marcel Henry s'est engagé en politique à partir de 1958 aux côtés de son oncle. Il participe à la fondation du Mouvement populaire mahorais (MPM) en 1963, parti favorable à l'appartenance de Mayotte à la France, dont il devient l'une des figures. Il est en effet l'un des plus ardents partisans du maintien de Mayotte dans la République. Il rassemble alors autour de lui de nombreux militants, notamment les « chatouilleuses », des femmes qui jouèrent un rôle décisif dans ce combat. Le 22 décembre 1974, la population de Mayotte se prononce à plus de 60 % pour le maintien dans la République, un amendement adopté par le Sénat lors du vote de la loi organisant une consultation des populations des Comores ayant permis un décompte des suffrages île par île. Le 8 février 1976, une nouvelle consultation est organisée à Mayotte, laquelle réunit 99,4 % des suffrages exprimés en faveur du maintien dans la République. Marcel Henry est élu sénateur en 1977. Lors de sa première intervention dans cet hémicycle, le 2 décembre 1977, il salue le rôle du Sénat en ces termes Les Mahorais savent le rôle éminent joué par le Parlement, et spécialement par la Haute Assemblée, dans la décision de la France de conserver Mayotte en son sein. Il affirme également : « En choisissant nettement, sans la moindre ambiguïté, de rester française, Mayotte a choisi la liberté. » À la suite de la consultation de 1976, la départementalisation devient le combat majeur de Marcel Henry.

La population mahoraise pense que cette première victoire [à savoir le maintien dans la République] doit être parachevée par l'accession au statut de département. Pour ma part, c'est la mission que j'ai reçue de ceux qui me font confiance depuis très longtemps et je ne m'en laisserai pas détourner. » Retiré de la vie politique à la fin de son mandat sénatorial participe cependant activement en 2009 à la campagne pour l'adoption du statut de département, proposé par le Président de la République Nicolas Sarkozy, laquelle aboutit le 31 mars 2011, date à laquelle Mayotte devient le cent unième département français. Au nom du Sénat tout entier, je souhaite exprimer notre sympathie et notre profonde compassion à la famille de Marcel Henry, à ses proches, à nos compatriotes mahorais,

L'ordre du jour appelle la discussion du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire dans les outre-mer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

Si je vous présente ces chiffres, c'est avant tout pour vous instruire de la situation de milliers de personnes infectées, en souffrance ou endeuillées, pour vous informer du combat que mènent les équipes médicales sur place, qui ne comptent ni leurs heures ni leurs forces pour sauver des vies vous rappeler l'esprit de solidarité qui anime les 2 000 soignants venus en renfort de leurs confrères antillais ou polynésiens depuis le mois de juillet. De cette tribune, je veux leur exprimer toute ma reconnaissance et leur dire un immense merci pour le combat qu'ils mènent pour et avec nos compatriotes d'outre-mer. La situation, dans certains territoires d'outre-mer, est dramatique. Il faut d'abord la regarder en face. Depuis le début de l'été, le Gouvernement et les services de l'État sont mobilisés pour protéger nos concitoyens ultramarins face à cette nouvelle vague.

l'état d'urgence sanitaire a été déclaré le 29 juillet, afin de mettre en oeuvre un couvre-feu et des mesures de confinement. Là encore, nous avons décidé de prolonger ces dispositions jusqu'au 19 septembre prochain. Le taux d'incidence en Guadeloupe reste extrêmement élevé- 520 cas pour 100 000 habitants. Les hôpitaux sont toujours soumis à une très forte pression 54 personnes sont actuellement hospitalisées en soins critiques, et le nombre d'admissions commence à peine à se stabiliser. À Saint-Martin et à Saint-Barthélemy, on constate une nette amélioration de la situation, qui permet au préfet délégué d'assouplir le couvre-feu.

L'état d'urgence y a été déclaré le 12 août dernier ; des mesures de couvre-feu et de confinement sont en vigueur. Au vu de la situation hospitalière, il est absolument indispensable de les maintenir.

Les mesures de freinage de la pandémie ont été renforcées dès le 20 août, avec notamment un confinement de la zone littorale, dite « zone rouge », où le virus sévit le plus sévèrement. À La Réunion, les mesures de freinage prises fin juillet commencent à porter leurs fruits, puisque les indicateurs Si le nombre de lits occupés par des patients atteints de la covid-19 diminue progressivement, une extrême vigilance reste néanmoins de mise. De premiers assouplissements progressifs

L'état d'urgence sanitaire a été déclaré hier par décret en conseil des ministres. La situation est d'autant plus alarmante que seuls 32 % des Calédoniens ont reçu au moins une dose L'Assemblée nationale a adopté mardi un amendement du Gouvernement tendant à préciser que l'état d'urgence sanitaire en Nouvelle-Calédonie s'appliquerait jusqu'au 15 novembre 2021, et ce avec l'accord de l'ensemble des formations et des forces politiques du Caillou, Je souhaite rappeler que, depuis le 1 juillet 2021, plus de 1 500 de nos compatriotes sont décédés à l'hôpital des suites de la covid-19 dans les outre-mer. Ce chiffre est glaçant ; il ne recouvre pourtant pas tous les décès, puisqu'il faut malheureusement y ajouter les personnes décédées à domicile. C'est pourquoi nous devons être capables de continuer à mobiliser tous les outils juridiques pour freiner la circulation du virus et stopper la saturation hospitalière. Sur ce plan, nous mesurons d'ores et déjà les effets des mesures de couvre-feu et de confinement. Il est donc impératif de les prolonger. Le projet de loi prévoit la prorogation de l'état d'urgence sanitaire

appelle une réponse immédiate et forte des autorités. La protection de nos compatriotes des îles Wallis et Futuna, qui partagent une bulle sanitaire avec la Nouvelle-Calédonie, s'inscrit dans cette logique, d'autant que le taux de vaccination y plafonne encore à un niveau trop faible.

Au total, près de 2 000 renforts humains ont été envoyés dans les outre-mer dans le cadre de cette quatrième vague. Des moyens matériels ont également été acheminés sans délai dans chaque territoire, y compris dans ceux où la santé ne relève plus de la compétence de l'État. en Polynésie française, outre des dizaines de milliers de tests, ce sont 32 concentrateurs d'oxygène et 50 000 blouses qui ont été acheminés. La solidarité nationale a également permis l'accueil de patients ultramarins, et notamment antillais, dans les hôpitaux de l'Hexagone.

Depuis le début de la crise, notre priorité est de protéger le tissu économique local en adaptant les outils de soutien aux besoins des territoires ultramarins. Nous continuerons en ce sens. Le fonds de solidarité est ainsi prolongé pour le mois de septembre dans les outre-mer. L'évolution de la situation sanitaire nous pousse en outre à en envisager le maintien au mois d'octobre.

les préfets referont un point complet avec les acteurs économiques. J'aurai l'occasion d'en rendre compte devant les deux assemblées. Le Gouvernement travaille aussi à un grand plan de reconquête et de transformation du tourisme. Les outre-mer y auront bien sûr toute leur place au regard de l'importance de ce secteur. Vous nous voyez

sur la situation des collectivités locales, car je sais le Sénat naturellement attentif à cet enjeu. Les filets de sécurité mis en place en 2020 pour le bloc communal et les régions ultramarines

Concernant les personnes décédées de la covid-19 dans les hôpitaux, 82 % n'étaient pas vaccinées. Je pèse mes mots en vous disant que l'adhésion à la vaccination rencontre plus de réticences- c'est le moins que l'on puisse dire -en outre-mer que dans l'Hexagone.

En Guyane, 25 % de la population totale a reçu une première injection et 19 % les deux injections. L'État ne ménage pas ses efforts de communication et a lancé des campagnes d'« aller vers » pour répondre à cet impératif sanitaire,

Comme à l'Assemblée nationale, j'appelle donc tous les responsables politiques et les personnalités de la société civile à se mobiliser en faveur de la vaccination. Désormais, prendre la parole, c'est sauver des vies.

au moment de prendre la parole à cette tribune, les premiers mots qui me viennent à l'esprit sont des mots de fraternité, de solidarité, d'émotion même,

l'unité politique, à la fois entre l'Assemblée nationale et le Sénat, et entre le Gouvernement et le Parlement, dans l'expression de cette profonde fraternité. Aujourd'hui, en effet, nous sommes tous Martiniquais, Guadeloupéens, Guyanais, Polynésiens ... Nous sommes tous Ultramarins. Nous avons tous une pensée pour nos compatriotes,

dont nous n'avions jamais fait l'expérience. En préparant cette intervention, j'avais à l'esprit le chiffre de 1 081

La situation de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Guyane, tout en n'ayant pas franchi le même seuil de gravité, est également extrêmement préoccupante, et même dramatique à certains égards. Il n'y a pas un outre-mer, mais des outre-mer. Il existe aussi des territoires qui, jusqu'à présent, ont été épargnés et qui ont su prévenir la propagation du virus par des mesures sévères. Je pense à la Nouvelle-Calédonie. Dimanche, je consultais nos collègues calédoniens : nous n'imaginions pas que, le Congrès de Nouvelle-Calédonie allait devoir prendre des mesures draconiennes de confinement. C'est dire s'il faut pouvoir s'adapter à l'évolution d'une réalité qui, malheureusement, parce que la France

Pour autant, il nous faut aussi parler des chiffres bien sûr. Vous l'avez fait, monsieur le ministre. Aussi n'y reviendrai-je pas trop longuement. On voit bien qu'il existe une corrélation

noter un frémissement pour la vaccination, et plus encore dans certaines collectivités. Plus les autorités sanitaires sauront s'appuyer sur des acteurs de confiance proches des habitants, ces derniers se reposeront sur une propagande indifférenciée, mieux cela vaudra. Les centres de vaccination éphémères et le recours aux médecins et aux infirmiers locaux constituent une démarche payante.

Il faut continuer, au-delà des mesures que nous pouvons autoriser en matière de confinement et de couvre-feu, l'effort de vaccination. La conviction, partagée par un nombre croissant de compatriotes d'outre-mer, que la vaccination les protège, protège leurs enfants et protège leurs parents, tel est le principal enjeu des semaines à venir.

les conditions d'habitat, la concentration des habitants dans des logements d'une dimension insuffisante pour éviter les contaminations, le taux de chômage, qui reste, dans certaines collectivités, trois à quatre fois supérieur à celui de l'Hexagone, montrent que rien n'arrive par hasard.

à prolonger l'état d'urgence sanitaire, là où il a déjà été décidé, jusqu'au 15 novembre, qui est la date d'échéance prévue par la loi sur le passe sanitaire. Je le propose aussi ; la commission a adopté cette disposition à l'unanimité. Cela ne veut pas dire que vous deviez absolument maintenir cet état d'urgence sanitaire jusqu'au 15 novembre Je me suis entretenu avec notre collègue de Saint-Barthélemy et j'ai échangé avec le président de cette collectivité. Il n'y a pas, aujourd'hui, de justification majeure à la pérennisation de l'état d'urgence sanitaire dans ce territoire. Je suis prêt à vous proposer, mes chers collègues, d'accepter que le Gouvernement puisse prendre cette décision de prolongation, mais je l'invite à réexaminer dans les prochains jours la situation de Saint-Barthélemy. Il ne faut pas que des collectivités subissent des contraintes qui ne sont que l'ombre portée des contraintes nécessaires dans d'autres collectivités, comme la Guadeloupe. La situation d'autres collectivités d'outre-mer mérite également un examen individuel très approfondi. Nous sommes tous étonnés de voir que Mayotte résiste à l'épidémie, et nous nous demandons si les chiffres qui nous sont donnés reflètent la réalité mahoraise. Je crains fort que les conditions ne soient réunies

les collectivités où vous demandez au Parlement d'autoriser, si vous deviez prendre un décret prononçant l'état d'urgence, que ce décret soit applicable non pas pendant trente jours, comme c'est normalement le cas depuis la loi du 23 mars 2020, mais jusqu'au 15 novembre prochain. Là aussi, sous bénéfice d'inventaire, je suis d'accord. Je l'ai dit tout à l'heure : pour la Nouvelle-Calédonie, nous pouvions encore nous interroger il y a quelques jours ; nous ne pouvons plus nous interroger aujourd'hui.

Pour que cette mesure soit pleinement efficace, il est nécessaire que les voyageurs se rendant en Nouvelle-Calédonie soient également vaccinés. Cette mesure relève d'un décret. Monsieur le ministre, peut-être pourrez-vous me répondre sur ce point. Avez-vous l'intention de de prendre ce décret dans les meilleurs délais ? Je n'ai pas cité toutes nos collectivités. Croyez bien, pourtant, que j'ai examiné leur situation particulière. notamment à Saint-Martin ; le partage de l'île entre la souveraineté néerlandaise et la souveraineté française, alors que les Pays-Bas n'appliquent aucune des règles que nous mettons en oeuvre, pose un problème pour l'efficacité des mesures, puisque la population circule sur toute l'île. Monsieur

de l'Assemblée nationale, pour lui demander d'exclure Saint-Pierre-et-Miquelon de la possibilité de prononcer un état d'urgence sanitaire de deux mois et demi, alors que le taux de vaccination y est nettement supérieur au taux hexagonal

ma contribution à la réflexion du Sénat sur la mise en échec de cette crise sanitaire dans nos outre-mer. Par ailleurs, je souhaiterais à mon tour m'associer à l'hommage qui a été rendu à notre ancien collègue Marcel Henry.

Monsieur le président, monsieur le président du Sénat, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous sommes d'abord ici pour exprimer notre solidarité à l'égard de nos compatriotes d'outre-mer frappés par une vague violente de ce virus aussi imprévisible qu'impitoyable, et pour saluer le magnifique élan de solidarité des soignants de métropole qui, par centaines, se succèdent en Martinique, en Guadeloupe et désormais en Polynésie, afin d'épauler leurs collègues, débordés par un flot de malades souvent dans un état très grave. Pour qu'une telle épreuve ne se cantonne pas à son côté désespérant, il faut en tirer les enseignements. Le premier d'entre eux- M. le ministre et M. le rapporteur l'on dit -, c'est le nombre démesuré des victimes dans les territoires peu vaccinés, alors que la métropole, grâce à un fort taux de vaccination, est en train d'éteindre la quatrième vague, après avoir contenu le nombre de cas graves. S'il fallait une preuve de ce que les scientifiques répètent depuis des mois, que le vaccin pour tous est la seule chance de vaincre le virus, cette preuve, nous l'avons sous les yeux, de la manière la plus éclatante et, malheureusement, la plus triste qui soit Cette preuve vient accabler, démasquer et dénoncer ceux qui depuis des mois tentent de discréditer le vaccin, d'effrayer les Français et de répandre leurs bobards sur des réseaux antisociaux devenus le fort Chabrol des agités du bocal et dans des cortèges de pigeons menés par des ânes, ces politiciens des deux extrêmes, dont les sermons vaccinosceptiques ne sont que le moyen d'atteindre l'objectif qui les obsède : foutre en l'air le système. Heureusement, comme dit le proverbe, le trot de l'âne ne dure pas longtemps. Après avoir jeté le soupçon sur le vaccin, forcé les autorités sanitaires à avancer à pas comptés et tenté de vider les vaccinodromes grâce à la désinformation, ils sont aujourd'hui pris à leur propre piège. Alors que les résistants d'opérette s'exprimaient dans les rues avec leurs pieds, tous les autres Français se sont exprimés avec leur cervelle en se faisant vacciner. Les Camille Desmoulins des boulevards de la démagogie avaient battu le rappel des antivax, des anti-système, des anti-Macron, des antisémites et surtout des « anti-tout les sondages leur révélant que même leurs propres sympathisants se partagent désormais entre antivax et vaccinés, ils tentent de sortir de la nasse en se mêlant au mouvement des anti-passe : je suis anti-passe, donc je ne suis pas vraiment antivax, je suis anti-passe donc je ne suis pas vraiment provax non plus. Avec ce double jeu, ils sont devenus la chauve-souris de la fable de La Fontaine : « Je suis Oiseau : voyez mes ailes [ ...] Je suis Souris ; vivent les Rats ». Heureusement, nous avons rarement vu une chauve-souris gagner l'élection présidentielle. Aujourd'hui, les cortèges ont fondu et les Français ont bien compris que la seule liberté que défendent ces leaders de pacotille, qui crient à la dictature en France tout en admirant Poutine et Maduro, est la liberté de mettre en danger la vie d'autrui au nom de théories qui tiennent plus du champignon hallucinogène que de la science et de certitudes acquises à l'université Facebook, section. Ils ne savent même pas localiser leur vésicule biliaire, mais ils ont un avis tranché sur l'ARN messager et l'hydroxychloroquine. Divine surprise ! Après un débat confisqué pendant des mois par des minorités aussi bruyantes que clairsemées, boursouflées par une couverture médiatique inversement proportionnelle à leur nombre, dans un drôle d'attelage à trois- les excités cherchant le bruit, les télévisions cherchant l'audience, les réseaux cherchant la haine -une majorité silencieuse de Français, de plus en plus solide, est montée en puissance pour défendre l'adhésion à des vérités rationnelles que les adeptes du glissement de terrain mental n'auraient jamais dû pouvoir mettre en doute. La décision courageuse des autorités de Nouvelle-Calédonie devant le risque terrifiant d'une nouvelle flambée nous montre aujourd'hui l'exemple. La vaccination obligatoire, ou en tout cas généralisée, est notre prochain défi. Les chiffres baissent partout, y compris aux Antilles. Sommes-nous à l'aube d'une victoire sur la pandémie ou n'est-ce qu'une simple trêve ? La réponse simple, claire et définitive à cette question est : « Dieu seul le sait. Le Gouvernement va devoir continuer à prendre des décisions délicates, difficiles, contestées par des irresponsables d'autant plus décidés à mettre le feu qu'ils viennent de subir une déroute. Faut-il décider d'une vaccination obligatoire en métropole ? Comment organiser les modalités de la troisième dose ? Comment maîtriser les risques à l'école, à l'université, dans les lieux publics ? Ce sont quelques-unes des questions que nous aurons à trancher ensemble dans les prochaines semaines, et le Sénat le fera avec le même sens de la responsabilité qu'il a su montrer jusqu'ici. Pour l'heure, il s'agit avant tout de parer au drame que vivent nos compatriotes d'outre-mer. Évidemment, nous voterons le projet de loi qui va le permettre.

l'interdépendance forte entre la santé des populations humaines et l'état de la biodiversité et des écosystèmes. Cette interdépendance est illustrée par le développement de nouvelles zoonoses

Ces chiffres diffèrent d'un territoire à l'autre et sont parfois éloignés de la réalité violente qui touche de nombreuses familles de nos concitoyens. Face à ce variant delta, le faible taux de couverture vaccinale est un facteur aggravant.

alors que, il n'y a pas si longtemps, ces mêmes autorités justifiaient, par exemple, l'utilisation du chlordécone uniquement pour les territoires de Guadeloupe et de Martinique, autorisation d'autant plus exceptionnelle que l'interdiction était en vigueur dans le reste du pays, à cause des effets néfastes reconnus de ce Les liens de confiance brisés sont les plus durs à réparer. Notre groupe appelle de ses voeux une meilleure communication : « l'aller vers », y compris, récemment, grâce à la possibilité donnée à tous les médecins commence par une information relayée à tous les niveaux par une diversité d'acteurs, dans un dialogue continu et soutenu, pour lever les peurs et les doutes. Ce constat de réticence n'est, nous le savons, pas seulement limité aux territoires d'outre-mer, mais à l'ensemble des territoires oubliés, voire abandonnés par la République, comme le montrent les écarts de couverture vaccinale récemment mis en avant, par exemple dans ma ville de Marseille. Comment Comment ne pas voir la similitude entre les zones à faible taux vaccinal et celles concentrant le plus de difficultés sociales et économiques et le plus de misère et de pauvreté ? Outre un taux vaccinal faible, ces territoires se trouvent particulièrement fragilisés : le système hospitalier y est vite saturé, malgré une mobilisation remarquable des personnels. Si l'hôpital va mal, si la diminution des moyens pour fonctionner et la fermeture de lits ont pesé ces dernières années et pèsent encore plus depuis le début de cette pandémie, cela est d'autant plus vrai dans ces territoires. Leurs structures hospitalières, de faible capacité, sont sous-équipées, et les évacuations sanitaires qui ont pu s'avérer nécessaires sont bien plus complexes et coûteuses qu'en métropole, en raison de leur isolement géographique. Ces mouvements de patients, comme ceux de médecins de soutien, sont l'exemple d'une solidarité nationale forte, mais qui ne saurait remédier durablement aux carences des politiques publiques. Mes chers collègues, il est important que le Gouvernement adapte la prorogation de la possibilité de déclarer l'état d'urgence en fonction des réalités de ces territoires si variés, et pourtant parfois traités comme un bloc homogène.

ne constitue en rien une obligation de prolongation jusqu'à cette date. Monsieur le ministre nous en a donné l'assurance, je l'en remercie. Aussi, notre groupe Écologiste- Solidarité et Territoires votera ce texte et apporte tout son soutien à nos concitoyens ultramarins. La

Monsieur le président, monsieur le président du Sénat, monsieur le ministre, mes chers collègues, Monsieur le ministre, les chiffres de la quatrième vague, que vous venez d'évoquer et qui frappe principalement la Martinique, la Polynésie française et la Guadeloupe, sont glaçants. Isolés les uns des autres, ils peinent pourtant à rendre compte de la réalité. Pour ne fournir qu'un seul exemple, puisque le temps m'est compté : entre le 20 et le 27 août dernier, douze personnes en moyenne sont décédées chaque jour de la covid-19 en Guadeloupe. Rapporté à la population française, cela représente le double de la moyenne nationale au plus fort de la première vague. C'est trop, beaucoup trop. Puisque l'occasion m'en est donnée, j'aimerais renouveler mon soutien ainsi que celui de mes collègues à l'ensemble des familles endeuillées, et aux malades qui parfois peinent à se rétablir. Permettez-moi également de saluer les soignants et l'ensemble des acteurs- collectivités, élus, bénévoles -qui oeuvrent sans relâche pour endiguer cette pandémie, et particulièrement ceux de l'Hexagone venus nous prêter main-forte et maintenir à flot nos hôpitaux sous tension. La situation sanitaire aux Antilles et en Polynésie française et la crainte de voir basculer le reste des territoires ultramarins

à y décréter, ou proroger, l'état d'urgence sanitaire. Nous le savons pourtant, ces mesures de court terme ne sauraient constituer une réponse satisfaisante à la crise. Les scientifiques nous le répètent, la vaccination reste à ce jour le moyen le plus efficace pour lutter contre l'épidémie de covid-19. Pour vacciner, au pays de Pasteur comme ailleurs, il faut d'abord rassurer. Il faut expliquer, et renforcer « l'aller vers » qui partout montre ses effets. En Guadeloupe, la région, le département et les communes s'y emploient depuis plusieurs semaines aux côtés de l'État. Un « vaccibus » a ainsi été affrété pour pallier un maillage territorial insuffisant des centres de vaccination. Il faut enfin s'attaquer à la désinformation qui, sur les réseaux sociaux notamment, détourne du vaccin, dans des proportions effrayantes, les plus indécis. Continuons donc de faire confiance à la science. La peur du vaccin et la méfiance à l'égard du personnel médical ne sauraient enfin justifier les menaces proférées à son encontre et les attaques dont il fait l'objet. Elles ne font que miner le moral et l'action de ceux qui nous protègent. Je terminerai brièvement en rappelant- et mon collègue Teva Rohfritsch complétera mon propos dans quelques instants -les difficultés que rencontrent l'ensemble des acteurs économiques de nos territoires, et particulièrement le secteur touristique et de l'événementiel. La prorogation de l'état d'urgence sanitaire doit en effet s'accompagner de mesures adaptées à un tissu économique constitué de très, très petites entreprises. Vous avez, monsieur le ministre, apporté à l'instant certaines précisions demandées par

Monsieur le président, monsieur le président du Sénat, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous sommes une fois de plus placés devant notre responsabilité de parlementaires afin de permettre, dans un cadre légal et proportionné, des mesures de protection exceptionnelles pour nos concitoyens d'outre-mer. L'urgence est là, sanitaire comme juridique. Cet été, la réalité d'un emballement du variant delta dans nos départements ultramarins a été criante. Les soignants nous ont fait part de leur désarroi face à l'afflux de patients, de leur crainte de devoir faire du tri, de leurs appels aux réservistes et, quand cela était possible, aux évacuations. Cette situation était d'autant plus choquante qu'elle faisait écho à la première vague vécue en métropole en mars 2020, durant laquelle nous ne disposions pas de vaccin. Mais elle était plus grave encore la contagiosité du variant, la prévalence de comorbidités, l'isolement insulaire, la capacité hospitalière et le faible taux de vaccination ont contribué à un état critique qui appelle la mobilisation de Compte tenu de la circulation très active du virus, le projet de loi tend à prolonger l'état d'urgence sanitaire jusqu'au 15 novembre 2021 en Guyane, à La Réunion, en Martinique, en Guadeloupe, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et en Polynésie Rappelons que la Guyane est en état d'urgence continu depuis le 17 octobre 2020, La Réunion et la Martinique depuis le 14 juillet 2021, la Guadeloupe, Saint-Barthélemy et Saint-Martin depuis le 29 juillet 2021, et la Polynésie française depuis le 12 août 2021. Les mesures concernant la Polynésie expirant le 11 septembre et celles concernant les autres territoires le 30 septembre, cette prolongation s'imposait, d'autant que l'école n'a pas repris partout.

Là encore, l'insécurité juridique, synonyme de recours, ne doit pas s'ajouter à une insécurité sanitaire. Aussi souscrivons-nous à cette stratégie qui protège les populations tout en assurant une certaine souplesse dans sa mise en oeuvre. Je souhaite ajouter quelques interrogations qui me paraissent déterminantes pour aider les Ultramarins à surmonter cette catastrophe sanitaire. Le conseil scientifique, dans son avis du 29 août, émet d'utiles recommandations pour adapter les politiques publiques.

Sur le plan scolaire- il n'est jamais trop tard pour s'en préoccuper -, comment la continuité pédagogique à distance est-elle assurée, sachant que les enfants ne peuvent aller à l'école et disposent dans certains cas de peu d'équipements ou d'infrastructures ?

les territoires d'outre-mer ont-ils des soignants et des structures adaptées pour prendre en charge les personnes atteintes de covid long ? Nous voterons en faveur de ce texte nécessaire et proportionné, tout en gardant à l'esprit que des politiques adaptées, visibles, structurelles permettront de redonner confiance à nos concitoyens et contribueront également à une meilleure protection sanitaire.

Les territoires ultramarins- donc celles et ceux qui y vivent et dont nous sommes solidaires -subissent les conséquences des politiques successives de sous-investissement dans les services publics et en particulier dans les services de santé, sous-dotés en soignants et en infrastructures. Cette situation a entraîné une explosion du nombre de malades de la covid-19 et une saturation des hôpitaux, notamment en Martinique et en Guadeloupe, marqués par un taux d'incidence excédant les 1 000 cas pour 100 000 habitants et un taux d'occupation des lits de réanimation supérieur à 96 %.

Face à cette situation, le Gouvernement demande au Parlement de proroger l'état d'urgence sanitaire en Guyane, en Guadeloupe et en Martinique et de l'étendre aux territoires de Saint-Pierre-et-Miquelon, de Mayotte, à la Nouvelle-Calédonie ainsi qu'à la Polynésie française. nous pensons qu'il est urgent d'accélérer la campagne de santé publique en faveur de la vaccination contre la covid-19 sans pour autant porter atteinte à nos libertés, une campagne qui ne stigmatise pas les populations pour leurs croyances, mais qui intègre clans son discours la domination de l'Hexagone et la méfiance à l'égard des organismes sanitaires perceptible depuis l'affaire du Mediator et, surtout, du chlordécone.

et des statistiques (Drees) sur les établissements de santé en France, la Guyane, la Martinique et la Guadeloupe sont les plus touchées par la sous-densité médicale, suivies en métropole par l'Île-de-France et le Centre-Val de Loire. Il s'agit donc d'une question d'égalité républicaine, mais également d'égalité sanitaire avec nos compatriotes ultramarins qui présentent des comorbidités spécifiques. Selon l'agence régionale de santé de Martinique, 95 % des patients admis en réanimation présentent au moins une comorbidité- hypertension, diabète, obésité, insuffisance respiratoire -et plus de 90 % des personnes hospitalisées sont en surpoids. La pandémie de covid-19 pointe les faiblesses de nos services publics, mais aussi les mesures urgentes à prendre. Face aux inégalités sociales de santé, le Gouvernement doit lancer un plan d'investissement en faveur des services de santé ultramarins, pour rattraper le retard accumulé depuis des années et répondre à d'éventuelles reprises épidémiques. L'article unique du projet de loi ne prévoit rien sur ce sujet et c'est fort regrettable. De la même manière, nous regrettons l'absence de comité de suivi associant les représentants de l'État, les professionnels de santé et les élus des territoires d'outre-mer. Le refus du Gouvernement d'accepter la proposition des parlementaires ultramarins qui veulent être mieux associés aux prises de décision n'est pas de nature à rétablir la confiance des populations à son L'annonce du Président de la République évoquant la possibilité de repousser la fin programmée du passe sanitaire et du régime de sortie de l'état d'urgence sanitaire après le 15 novembre pose également question. Le Gouvernement envisage-t-il de repousser l'état d'urgence sanitaire au 28 février, date de fin de la session parlementaire, ou jusqu'au 30 juin, c'est-à-dire après les élections, présidentielle et législatives ? La perspective de l'organisation d'une campagne électorale présidentielle et législative sous état d'urgence sanitaire n'est pas acceptable pour nous. En conclusion, les sénatrices et sénateurs du groupe CRCE voteront contre ce projet de loi qui porte atteinte aux prérogatives du Parlement et réduit les libertés publiques de manière disproportionnée, en cohérence avec leurs votes sur les précédents projets de loi portant sur l'état d'urgence. La parole est

La situation sanitaire des outre-mer s'est considérablement dégradée depuis quelques semaines en raison de la propagation spectaculaire du variant delta de la covid-19. Je voudrais exprimer notre solidarité et notre fraternité envers nos compatriotes de ces différents territoires. C'est tout particulièrement le cas chez moi, en Polynésie, où nous déplorons le décès de plus de 535 personnes.

En matière de taux de vaccination, d'énormes efforts sont réalisés par l'ensemble des instances locales pour accélérer la campagne et atteindre notre objectif. Plus de 144 000 Polynésiens ont reçu la première dose et plus de 120 000 ont un schéma vaccinal complet, sur un nombre total de 276 000 habitants.

par ambulance, par avion, par hélicoptère et parfois même par bateau, quand l'île ne dispose pas de piste d'aviation. Ces difficultés, liées à notre spécificité géographique, ne se retrouvent nulle part ailleurs.

La solidarité nationale a aussi pleinement joué son rôle, par l'envoi de renforts sanitaires et de matériels médicaux. Permettez-moi, à ce titre, de remercier le ministre des solidarités et de la santé, le ministre des outre-mer, le président du Sénat ainsi que toute la représentation nationale. Depuis plusieurs semaines, un couvre-feu a été établi en Polynésie et les îles des archipels les plus touchés sont confinées depuis le 23 août 2021. Cette situation de crise sanitaire provoque évidemment une crise économique et financière d'une très forte ampleur, qui se traduit par une baisse de plus de 12 % du PIB, et la perte de nombreux emplois.

La collectivité a dû faire face à cette situation. Le pays a ainsi supporté pas moins de 73 457 246 euros de dépenses

relatives aux dispositifs d'aide au maintien des emplois, ou encore les dépenses de l'Institut Louis-Malardé et les pertes constatées de notre compagnie aérienne. Lorsque le Président de la République s'est rendu en Polynésie française, il a témoigné avec force de la solidarité de l'État envers notre collectivité et a pris quelques engagements. J'en retiens en particulier trois. de développement (AFD) d'un prêt de 300 millions d'euros garanti par l'État afin de financer la crise, mais aussi, et surtout, la relance de l'économie polynésienne. Il est important que les instances de l'AFD puissent accorder ce concours, puis procéder à la signature de la convention qui s'y rapporte. De même, la prochaine loi de finances rectificative doit expressément prévoir la garantie de l'État. la République concerne le soutien de l'État à la compagnie aérienne locale Air Tahiti Nui. Il faut que l'État puisse aider l'ensemble des transporteurs ultramarins de manière équitable. le troisième sujet concerne le maintien des dispositifs d'aide en faveur des entreprises. M. le ministre de l'économie et des finances a annoncé que les dispositifs du fonds de solidarité de l'État seraient reconduits jusqu'à la fin de l'année. C'est une très bonne décision, dont je sais qu'elle sera appréciée par les professionnels concernés en outre-mer. Ainsi, compte tenu de la situation sanitaire qui prévaut dans les outre-mer, il est évident qu'il convient de proroger l'état d'urgence sanitaire décrété depuis le 11 août. la mise en oeuvre des mesures destinées à lutter contre l'épidémie pose une réelle et grave difficulté pour les collectivités du Pacifique. En effet, il appartient désormais exclusivement aux autorités de l'État de prendre toutes les mesures nécessaires sur le territoire de la Polynésie française, et ce nonobstant le partage des compétences établi par la loi organique statutaire du 27 février 2004 qui confère à la collectivité d'outre-mer la compétence de principe et à l'État une compétence d'exception. Ainsi, la proclamation de l'état d'urgence sanitaire a eu pour effet de réduire à néant certaines compétences de la Polynésie française, désormais exercées par l'État. En temps « normal », où prévaut en principe le droit commun, la Polynésie française est compétente en matière de santé publique et dispose aussi du pouvoir de police administrative en matière sanitaire, ce qui lui permet de lutter contre les fléaux dont pourraient souffrir les Polynésiens. Mais, en raison de la proclamation de l'état d'urgence sanitaire due à cette période exceptionnelle, et qui tend, hélas ! à devenir le droit commun, les compétences de la Polynésie doivent s'effacer au profit de celles de l'État, et plus particulièrement du haut-commissaire Ce nouvel état du droit pose deux problèmes. Tout d'abord, il ne me semble pas totalement conforme à la jurisprudence du Conseil d'État, puisque la Haute Assemblée, dans un avis du 15 mars 2005 relatif à la sécurité et à la sûreté en matière aérienne, a considéré qu'« il appartient à l'État de financer les missions qui lui incombent sur le territoire » de la collectivité de Polynésie française. Aussi, il convient de se demander s'il n'appartient pas à l'État de supporter les charges relatives à la lutte contre la pandémie, qui, pour l'instant, incombent exclusivement à la Polynésie française. Ensuite, ce nouvel état du droit instaure, d'une certaine manière, une forme de « curatelle » pour les collectivités d'outre-mer dotées de l'autonomie, ainsi que pour la Nouvelle-Calédonie. de mettre fin à cette situation de mise sous tutelle, qui a des relents d'un passé révolu ? Autrement dit, la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie ne devraient pas être censurées en termes de compétences, mais sur le plan de la légalité interne. Certes, Certes, il s'agit là d'un autre débat qui touche à l'évolution statutaire. Cependant, dans un proche avenir, il faudra envisager une réforme statutaire des collectivités d'outre-mer. Le groupe Union Centriste votera ce texte. La parole

Monsieur le président, monsieur le président du Sénat, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous examinons aujourd'hui un texte simple, technique, globalisant, à harmoniser la réponse apportée à la quasi-totalité des territoires et collectivités des outre-mer, y compris désormais la Nouvelle-Calédonie. C'est justement en Nouvelle-Calédonie, territoire longtemps épargné, que, dans un élan transpartisan et dans un souci supérieur de protection, les élus viennent de décider à l'unanimité d'instaurer l'obligation vaccinale- décision remarquable et exceptionnellement courageuse.

que ce texte seul ne sera pas suffisant. Soyons clairs : cela fait maintenant plusieurs semaines que nous avons dépassé le simple stade de l'état d'urgence ; nous faisons bel et bien face à une catastrophe sanitaire, sociale et humanitaire. relève désormais d'une médecine de guerre, la pandémie ayant fait imploser nos systèmes de soins. Impuissants, nous avons vu l'opinion et nos familles se déchirer ; impuissants, nous comptons désormais nos morts. Pour ne plus pleurer et subir, pour ne plus improviser et brusquer, il s'agit maintenant de comprendre pourquoi et comment nous en sommes arrivés là, pour éviter, autant que faire se peut, une répétition de ce drame. Malgré trois vagues successives en moins d'un an, il y a eu manifestement carence fautive d'action- et peut-être de pensée -et défaut cruel d'anticipation de cette quatrième vague. Nous savions en effet que, pour ces populations, les nôtres, « vaccinées » douloureusement par l'Histoire, la résistance et la méfiance séculaire contre toutes les paroles d'autorité- et singulièrement celle de l'État -seraient un obstacle considérable à la vaccination. Citoyens disciplinés, nous avons accepté les confinements, supporté les couvre-feux, compris les nécessaires restrictions de libertés. Mais comment a-t-on pu laisser les réseaux sociaux s'emparer de manière aussi obsessionnelle des esprits et imposer une pensée obscurantiste ? Comment peut-on encore lire, sans riposte claire et convaincante, que le vaccin est dangereux ? Comment justifier ce manque de lits de réanimation, ce manque de personnels, ce manque d'oxygène, ce manque criant d'eau, ce manque de seringues, de cathéters, de sondes de respiration, ce manque de centres permanents de vaccination, de linge et de gants, de « vaccibus ce manque de pédagogie et de proximité dans la stratégie vaccinale ? Comment comprendre cette communication détachée des caractéristiques culturelles de ces peuples, de leurs croyances, de leur histoire ? Dès le mois de mai, nous savions que ce cocktail risquait d'être explosif. Il est devenu meurtrier, terriblement meurtrier. En disant cela, j'ai l'honnêteté de reconnaître, monsieur le ministre, que le Gouvernement a agi. Je soutiens cet effort, mais si je n'ignore rien, vous l'aurez compris, je ne vous exonère de rien non plus. Sur des territoires déjà sous-dotés, fracturés et gangrenés par la misère, votre manque d'anticipation et de projection a, en partie, amplifié les effets de cette crise. Si, comme chacun ici, je salue et remercie les personnels soignants pour leur dévouement sans faille, malgré leur épuisement moral, psychique et physique, je dis aussi de la santé ne pourra, demain, constituer la seule réponse des autorités. Je continue donc de demander une refonte globale de la politique sanitaire outre-mer. Je plaide pour plus d'anticipation et donc de moyens. Je plaide aussi pour une plus grande capacité de projection pour affronter une possible cinquième vague, en moyens, en proximité, en personnels, en équipements et en véritable démocratie sanitaire. en effet à la fois blessant et injuste de faire porter cet échec sur la seule résistance aux vaccins : cette vague n'est pas entrée par effraction dans nos vies, elle est aussi la conséquence d'un sous-investissement chronique dans notre système de soins. Socialistes, nous croyons à la science, à la médecine et au progrès. Forts de la double éthique de conviction et de responsabilité qui est la nôtre, nous persistons à dire que la vaccination obligatoire reste, à cette heure, la seule voie pour sauver des vies, sauver des vies, préserver la liberté de tous, garantir la protection de chacun et assurer un retour à la vie normale. Bien sûr, je comprends les doutes, les craintes et les peurs. Bien sûr, je mesure et je n'ignore pas les traumatismes de contaminations gravés dans la mémoire collective, mais face aux milliers de morts, j'estime avoir le devoir moral et humain de tout faire pour contribuer à sauver des vies et mieux nous armer pour affronter la cinquième vague. Face aux réticences et aux oppositions, face à la peur et à la désinformation, votre stratégie doit manifestement évoluer, car elle a parfois nourri la méfiance et la dissonance. Aimer, c'est aussi protéger. Je vous demande donc de repenser profondément votre politique sanitaire dans les outre-mer.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, je n'appartiens pas à la majorité gouvernementale- je siège, comme vous le savez, dans l'opposition -, mais je pense que, face à la gravité

que la Martinique et La Réunion ont reconfiné à la fin du mois de juillet, suivies de près par la Guadeloupe au début du mois d'août. Le territoire de Saint-Martin subit des restrictions quasiment en continu depuis le début de la crise. la vaccination et l'immunité collective reste un objectif difficile à atteindre du fait de la partition de l'île. Le grand nombre de contaminations a provoqué des tensions au sein du centre hospitalier Louis-Constant Fleming, qui ne dispose que de très peu de places, pour près de 40 000 habitants. Si la situation est alarmante, c'est aussi en raison de la faiblesse de nos moyens hospitaliers. Certes, le nombre de contaminations baisse grâce aux mesures de confinement, mais trop faiblement. La situation reste inquiétante, car les seules marges de manoeuvre dont nous disposons sont le transfert de patients chez nos voisins guadeloupéens ou martiniquais, eux-mêmes sous tension.

nous avons tous des proches frappés par cette épidémie. À cet égard, je tiens à adresser ici mes pensées les plus sincères et solidaires à la population saint-martinoise, ainsi qu'à tous les personnels de santé, qui s'épuisent pour soigner les nôtres. Si j'entends quotidiennement l'expression d'une détresse profonde, je reçois également des propositions constructives de mon territoire, qui méritent d'être écoutées et discutées. Il ne saurait y avoir d'état d'urgence sanitaire- de surcroît prolongé -sans mesures d'accompagnement tout aussi urgentes, davantage adaptées à nos territoires. Le Gouvernement y a déjà en partie répondu par des mesures de soutien spécifiques à nos économies et je l'en remercie. Ces mesures doivent être le pendant naturel de la prolongation de l'état d'urgence sanitaire. Par ailleurs, permettez-moi de vous rappeler, monsieur le ministre, que Saint-Martin connaît une situation particulière du fait de sa partition : une vaccination du côté français sans concertation avec le côté néerlandais risque de réduire fortement l'efficacité de la vaccination sur la population. J'attire également votre attention sur les difficultés que poserait une éventuelle mise en place d'un passe sanitaire sur la seule partie française de l'île. Elle ne manquerait pas de provoquer des complications pour notre territoire. l'asymétrie des conditions d'accès à l'île. Saint-Martin est une destination touristique dont les infrastructures internationales d'accueil, port et aéroport, sont installées dans la partie néerlandaise, où le passe sanitaire n'existe pas. De surcroît, les comportements de consommation sur l'île se feront encore plus au détriment des commerces, restaurants ou autres lieux d'activités de la partie française. La libre circulation des biens et des personnes restant le principe à Saint-Martin,

qui ne manqueront pas de peser sur l'ensemble de l'industrie touristique de l'île, laquelle est vitale pour notre économie, notre population et notre territoire tout entier. Il en est de même pour la fixation des horaires de confinement. Comment comprendre que la partie française soit soumise à un horaire différent de la partie néerlandaise ? C'est pourquoi une concertation avec le gouvernement de Sint Maarten me semble absolument indispensable, afin notamment de mettre en place des protocoles sanitaires communs, voire de mutualiser les moyens locaux et étatiques. Au regard de la situation spécifique du territoire, il me paraît urgent d'envisager rapidement la tenue d'un comité regroupant les gouvernements français et néerlandais, la collectivité de Saint-Martin et le gouvernement de Sint Maarten, dans le cadre d'un « Q4 sanitaire Je souhaite avoir votre sentiment sur ce point, monsieur le ministre. La parole Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, la Polynésie française est en deuil ; la Guadeloupe, la Martinique également Saint-Barthélemy, Saint-Martin, la Guyane et La Réunion n'ont pas été épargnées. À peu d'exceptions près, nos territoires ultramarins sont tous en alerte. Même nos amis et voisins calédoniens ont détecté récemment des cas de covid-19 parmi la En Polynésie, on décompte 44 000 cas dépistés positifs en cumul sur 277 000 habitants. Le taux d'incidence est monté fin août à plus de 3 500, à 4 000 aux îles Sous-le-Vent. C'est dramatique pour les malades, car tous n'accèdent pas aux soins dont ils ont besoin ; c'est terrible pour les soignants, qui sont à bout de forces et condamnés à faire des choix angoissants pour nos familles. Nous avons passé ce week-end la barre des 513 morts. Ces chiffres peuvent paraître relativement faibles à l'échelle de la Nation.

En outre-mer, nous faisons face avec gravité à notre vulnérabilité, à notre éloignement, mais aussi à l'état de santé de nos populations, aux maladies non transmissibles, sans oublier les difficultés liées à l'habitat insalubre ou indigne, à la promiscuité pour de trop nombreuses familles. vaccination est un facteur aggravant. Nous vivons un drame, non pas ultramarin, mais national. Nous devons, là-bas comme ici, en tirer les leçons. C'est aussi dans de pareils moments que nous devons être plus forts tous ensemble, solidaires au sein de la République, solidaires entre Français.

Merci aussi à tous nos amis calédoniens pour leur aide précieuse en renfort dès les premiers temps. Merci enfin de réunir le Parlement pour prolonger les outils législatifs nécessaires pour stopper les chaînes de contamination. Oui, la vaccination a enfin fait un bond en Polynésie, certainement dopée par la dure réalité de la mort. Les et autres doctorants des réseaux sociaux ont mis à mal les campagnes de vaccination. Certaines obédiences religieuses ont aussi chez nous une lourde responsabilité. « Aller vers », convaincre, rassurer et vacciner restent aujourd'hui plus que jamais les priorités de tous. Nous ne devons rien lâcher de ce point

Nous connaissions déjà les cyclones dévastateurs, nous voici désormais en proie aux épidémies meurtrières. Nos géographies ne sont pas des boucliers, elles sont au contraire un risque supplémentaire. Nous devons collectivement réfléchir aux moyens de garantir à tous nos citoyens un socle commun de prise en charge sanitaire adapté à cette nouvelle donne internationale. C'est non pas une question de statut ou d'« ultramarinité », mais de priorité et de moyens consacrés à la santé des Français. Nous l'évoquerons certainement lors du prochain débat budgétaire : nos économies locales souffrent également. : nos économies locales souffrent également. La santé, la vie des Français sur chacun des océans qui composent la République restent les priorités du jour. Merci, chers collègues de voter avec nous en faveur de ce projet de loi.

soutenir une industrie incapable de résister à une concurrence effrénée. Ce sont ces dérogations que j'aurais pu solliciter pour donner les moyens à ce magnifique pays de s'inscrire résolument dans l'espérance. Mais, hélas, entre espoirs perdus et désillusions, la réalité est tout autre.

faute de soins, faute de médecins ! Nos hôpitaux, déjà fragiles, se sont trouvés submergés, malgré les renforts et les moyens déployés pour faire face à la crise. Nos soignants, auxquels je rends hommage, sont à bout de souffle. Et personne ne peut dire aujourd'hui quand viendra le moment du répit

Une île ne peut pas compter sur les départements voisins en cas de problème. Il est donc désormais impératif de faire vite pour consolider nos hôpitaux, prendre des mesures afin de faciliter l'implantation de nouveaux médecins et revoir nos capacités d'accueil en réanimation. Nous voterons, par nécessité, la prorogation de l'état d'urgence sanitaire. Nous la voterons, car la gravité de la situation ne nous laisse pas d'autre choix. Il faudra cependant -nous assumions courageusement nos responsabilités. Je ne suis pas du genre à les rechercher uniquement chez les autres : notre crédulité face à cette pandémie, une certaine frilosité ambiante locale quant à la nécessaire

Il nous faut désormais faire plus pour convaincre jour après jour et rassurer des populations qui doutent face au vaccin. Il faut amplifier la stratégie vaccinale de proximité et aller encore plus vers les gens, ceux qui ne peuvent pas se déplacer, ceux qui sont éloignés de tout. En effet, à ce jour- désolée de le dire, mais je l'assume -, nous n'avons pas de solution plus efficace que le vaccin contre les formes graves de la maladie. Dans le même temps, nous devons aussi évoquer la question de nos entreprises,

aujourd'hui, de nombreuses entreprises n'y ont pas accès. Il faut faciliter la mise en place de plans d'apurement des dettes sociales et fiscales de nos sociétés et, surtout, raccourcir les délais d'instruction. Des mesures devront être prises pour limiter l'impact social d'une crise dont l'ampleur nous inquiète. Pour finir, je voudrais parler d'éducation. En Martinique, les écoles sont restées fermées de façon quasiment continue de décembre 2019 à septembre 2020, et la continuité pédagogique a été très inégale. Le confinement a de nouveau contraint notre académie, comme celles d'autres

à l'arrivée en CE2, un élève sur deux ne sait pas déchiffrer les lettres ! Un plan ambitieux pour l'éducation sera nécessaire. Nous ne pouvons pas laisser nos enfants être les grands sacrifiés du covid.

nous entamons les travaux parlementaires de septembre par un nouveau texte consacré à la crise sanitaire qui frappe malheureusement depuis maintenant plus d'un an le monde entier. Les Français de l'Hexagone en ont évidemment fait l'expérience, mais il faut se garder d'oublier que le tempo de l'épidémie n'est pas le même partout dans le monde : les Français de l'étranger, que j'ai l'honneur de représenter, peuvent en attester. Il en est de même pour nos compatriotes ultramarins, dont il est question aujourd'hui. Je ne reviendrai pas en détail sur des situations particulièrement difficiles parfois, dont nos collègues représentant les différentes collectivités d'outre-mer se sont fait l'écho. Il est incontestable que les mois de juillet et d'août se sont révélés singulièrement éprouvants, en particulier dans les départements et territoires des Antilles, en Guyane, mais aussi, plus récemment encore, en Polynésie française. En ces heures difficiles, nos pensées et notre soutien vont bien évidemment aux habitants des outre-mer, en particulier aux familles endeuillées et aux soignants. Les causes de cette dégradation soudaine des situations sanitaires locales sont nombreuses et complexes. Elles sont souvent liées aux vulnérabilités structurelles nées de capacités hospitalières limitées et d'une isolation géographique compliquant le transfert de patients. À cela s'ajoutent des taux de vaccination souvent significativement plus faibles qu'en métropole. Or, comme notre rapporteur l'a relevé, le taux d'incidence du virus est souvent le plus élevé là où le taux de vaccination est le plus bas. Confronté à cette situation, le Gouvernement a fait le choix de demander au Parlement la prorogation de l'état d'urgence sanitaire dans plusieurs de ces collectivités ultramarines. L'article 3 de la loi du 31 mai 2021 prévoyait en effet que cet état d'urgence devait perdurer jusqu'au 30 septembre 2021. Pis, la Polynésie française a depuis lors fait face à un pic épidémique : les taux d'incidence épidémique : les taux d'incidence sont supérieurs à 3 000 dans certains archipels. Logiquement, le Gouvernement y a déclaré l'état d'urgence sanitaire par décret le 11 août. Mais cet état d'urgence sanitaire, qui ne peut durer plus d'un mois sans intervention du législateur, arrive désormais à son terme. Compte tenu des conditions actuelles sur le terrain, conserver ces dates de fin d'état d'urgence sanitaire dans les outre-mer n'était pas réaliste. La commission des lois a dès lors accueilli favorablement la prorogation de ces dispositifs jusqu'au 15 novembre,

Les travaux des derniers jours ont aussi permis d'ajuster le projet de loi initial. C'est ainsi que les discussions entre les rapporteurs de l'Assemblée nationale et du Sénat ont abouti au retrait de Saint-Pierre-et-Miquelon du texte, cette collectivité combinant faible incidence et haut taux de vaccination. Les récents développements en Nouvelle-Calédonie ont également conduit à l'adoption, par les députés, d'une disposition introduisant ce territoire dans le texte, ainsi que les îles Wallis et Futuna. Si ces collectivités ont jusqu'ici évité le pire, il demeure crucial de prendre en amont des mesures de freinage du virus et d'épauler le gouvernement calédonien dans la gestion de la situation. Par ailleurs, ce qui est valable pour la Nouvelle-Calédonie peut aussi l'être pour les autres collectivités. Certes, nous nous apprêtons à voter la prorogation de l'état d'urgence sanitaire, dans certains cas par anticipation, mais cela n'implique pas que celui-ci doive s'imposer de manière uniforme partout, ni jusqu'au 15 novembre. Au contraire, nous incitons l'exécutif au dialogue avec les différentes collectivités ultramarines afin d'adapter les mesures prises à la situation de chaque territoire et, le cas échéant, de mettre un terme à l'état d'urgence là où il pourrait ne plus être nécessaire. Au moment où les outre-mer sont dans une grande détresse du fait de l'épidémie, la solidarité nationale et le dialogue sont plus que jamais de mise. Vous l'aurez compris, le groupe Les Républicains, en phase avec la position du rapporteur, votera ce texte et appelle de ses voeux un vote conforme et une promulgation rapide de la loi. Très bien

Soyons bien clairs, une coordination a lieu en permanence à l'échelle locale entre le préfet délégué et les autorités de Sint Maarten. Pour être honnête, je me dois de dire que, si les différentes interventions de la République, de l'État, des autorités diplomatiques vis-à-vis du royaume batave produisent des effets, Sint

Il est clair que nous coordonnons tout ce que nous pouvons coordonner, jusqu'au moment où les autorités de l'autre côté de la frontière ne souhaitent pas le faire ou ne veulent pas s'aligner sur ce que nous proposons.

de stratégies hospitalières et de santé publique beaucoup plus adaptées aux territoires d'outre-mer. Une agence régionale de santé a-t-elle vocation à fonctionner de la même manière dans un territoire monodépartemental tel qu'une île

qui permettent aux autorités sanitaires, d'une part, et aux préfets, d'autre part, d'associer le monde médical, public comme privé- y compris d'ailleurs les pharmaciens, qui ont un rôle encore plus particulier en outre-mer que dans l'Hexagone -, et l'ensemble des élus locaux. J'ai entendu à l'Assemblée nationale la même

Enfin, se pose la question des compétences. Elle est très importante, car elle renvoie à la Nouvelle-Calédonie et intéresse l'ensemble des parlementaires qui se passionnent pour ces sujets.

En revanche, madame la sénatrice, il n'est pas exact de dire que l'état d'urgence sanitaire écrase les compétences de la Polynésie. En tant que pays, la Polynésie est, en droit,

vers », nous n'en sommes pas là ... La sénatrice Conconne peut en parler, elle qui s'est mobilisée. On a malheureusement affaire à des groupes qui allient désinformation et récupération politique. Les réseaux sociaux,

d'autres connexions avec l'Hexagone, pour les raisons que vous connaissez. Autant de sujets sur lesquels nous devrons évidemment nous pencher ... Pardonnez-moi, monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, j'ai été un peu long, mais je souhaitais apporter les réponses les plus précises possible à l'ensemble des questions qui m'ont été posées.

et de la Martinique. Il y a également des surcoûts exorbitants dans nos territoires, et je souhaiterais vraiment que vous preniez en compte les coefficients géographiques que j'ai souvent évoqués dans mes amendements.

Comme je l'ai évoqué précédemment dans la discussion générale, la Polynésie traverse actuellement une période difficile, particulièrement au niveau sanitaire, et inédite en termes de décès enregistrés à ce jour. jour. alors de nos us et coutumes totalement mis à mal, car nos familles ne peuvent plus réellement faire le deuil de leurs chers disparus ? La meilleure décision que nous aurions dû prendre pour éviter cette catastrophe humaine était la fermeture de nos frontières, avec un confinement général sur l'ensemble du territoire. Mais tel ne fut pas notre choix, et nous l'assumons, car les stigmates des précédents confinements restent encore visibles, au plan tant social qu'économique. La gestion de cette crise depuis mars 2020 a aussi mis en exergue une mise sous tutelle de certaines de nos compétences. Par moments, nous avons eu l'impression que l'État décidait de tout. Et ce n'est pas l'élue derrière un écran qui vous parle,

Karoutchi -nous demandons que le Gouvernement s'engage à faire inscrire dans la prochaine loi de finances pour 2022 une contribution exceptionnelle contribution exceptionnelle pour venir compenser les pertes de recettes et les dépenses engagées sur l'exercice 2021 par la Polynésie pour la gestion de cette crise. Nous étions prêts à déposer un amendement pour illustrer nos propos, mais, en parfaite cohérence avec la commission des lois du Sénat et de l'Assemblée nationale pour aboutir à un vote conforme, nous ne l'avons pas fait. C'est ainsi que je demande avec force et conviction au président du Sénat

Philippe Bas. Déjà, en juillet dernier, lors du neuvième texte sur l'état d'urgence, les spécificités des territoires avaient été relevées, notamment par notre rapporteur Chantal Deseyne. La situation était déjà tendue.

s'attaquer » à ce sujet spécifique, en partenariat avec nos collègues de la commission Annick Petrus, Dominique Théophile, Victoire Jasmin et, bien entendu, le président de la délégation sénatoriale aux outre-mer, notre collègue de Saint-Pierre-et-Miquelon Stéphane Artano.

nous ! La parole est à M. Dominique Théophile, sur l'article. Permettez-moi, par le biais de ce texte, d'appeler votre attention sur deux sujets que nous devons garder à l'esprit, à l'heure où nous prolongeons l'état d'urgence sanitaire pour protéger les populations. Tout d'abord, la crise sanitaire a joué un rôle de catalyseur des problèmes de santé mentale, mettant en exergue la nécessité de porter une attention spécifique à cette dimension. Les décisions prises pour freiner l'épidémie comme les confinements ou l'incitation au télétravail bouleversent le quotidien et les relations sociales personnelles comme professionnelles, avec des conséquences diverses sur la santé mentale. La dépression ou l'anxiété sont des pathologies qui sont de plus en plus diagnostiquées, comme en témoignent les principaux indicateurs de santé mentale analysés par Santé publique France. En 2019 déjà, l'enquête santé européenne indiquait que le taux de symptômes dépressifs et de symptômes dépressifs majeurs était significativement plus élevé en outre-mer qu'en métropole. Il nous reviendra d'intégrer les conséquences de la crise sur la santé mentale des Ultramarins au lourd bilan de cette épidémie et d'y apporter des solutions adéquates, avec une meilleure prise en compte des besoins, une meilleure répartition des professionnels de santé mentale vers les lieux de vie et un suivi plus assidu des pathologies. La crise sanitaire a également démultiplié les situations de précarité dans l'Hexagone. Les ménages vulnérables en outre-mer ne sont pas épargnés. Ils se retrouvent dans une grande précarité. Nous devons aussi les soutenir, les accompagner et nous montrer solidaires, dans l'esprit du « et

Cohen, sur l'article. J'apprécie l'intervention de Catherine Deroche, mais je m'étonne quelque peu. Elle ne peut pas parler au nom de la commission, qui n'a pas été saisie pour avis, ce que je regrette profondément.